Merci,

soir. La problématique du Grand Paris n'est pas nouvelle. Dès le XIX siècle, deux visions se sont opposées : celle de Napoléon III, ... Eh oui ! ... qui imaginait une capitale s'étendant de Saint-Germain-en-Laye à Marne-la-Vallée, Marne-la-Vallée, s'est heurtée au réalisme du baron Haussmann, qui a fait justement remarquer qu'il avait fallu un combat de dix-sept ans pour unifier l'ensemble des communes d'Auteuil, de Passy ou des Batignolles et créer la ville de Paris.

Il indique que tout reste à faire pour répondre aux nombreux problèmes de l'agglomération parisienne : inégalités territoriales, logements, transports, services publics ... En 1949, le célèbre géographe Jean-François Gravier, auteur de, propose la création de seize régions avec des superpréfets ainsi que d'un « Grand Paris ». Toutefois, la réforme de l'Île-de-France organisée par la loi du 10 juillet 1964 a eu raison de cette vision. Les trois départements créés en 1790- Paris, la Seine-et-Oise et la Seine-et-Marne -sont subdivisés en sept nouveaux départements : la petite couronne et la grande couronne. couronne. La réorganisation de l'Île-de-France redevient un sujet de conversation au début des années 2000, face au constat partagé d'un développement économique déséquilibré : pas de desserte ferroviaire directe entre le centre de Paris et ses aéroports ; difficultés à rejoindre le pôle technologique de Saclay

C'est la loi de juin 2010, relative au Grand Paris, qui définit ce territoire comme « un projet urbain, social et économique d'intérêt national

Marseille. En première lecture, le Sénat rejette l'ensemble des articles relatifs à la zone parisienne. C'est l'Assemblée nationale qui dessine ce qui sera plus tard la métropole du Grand Paris, la MGP. En septembre 2013,

L'opposition des élus s'est renforcée après les élections municipales de 2014, lesquelles ont modifié l'équilibre au sein du territoire métropolitain. à l'unanimité, les élus de Paris Métropole réclament une révision de l'article 12 de la loi Maptam, qui supprime les intercommunalités. Cette position est réaffirmée quelques mois plus tard en octobre 2014, quelque 94 % des membres de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris réclament une personnalité juridique pour les territoires et un partage des recettes de la fiscalité économique.

Sur les 11 territoires créés au sein de ce périmètre, seuls 3 préexistaient ; les 8 autres ont été imposés par les préfets et font parfois l'objet de mariages forcés. Non soutenue par les maires, cette nouvelle organisation est restée un échelon supplémentaire dans une organisation territoriale déjà très compliquée, comprenant communes, territoires, départements, métropole, grands syndicats et région. Chacun cherche à conserver les compétences que la loi lui a retirées. À titre d'exemple, une seule opération d'aménagement, la zone d'aménagement concerté, ou ZAC, des docks de Saint-Ouen, a été transférée à la métropole du Grand Paris lors de sa création. Seuls deux actes ont depuis été déclarés d'intérêt métropolitain. Par ailleurs, la MGP reste un nain budgétaire. Si elle enregistre 3,4 milliards d'euros de ressources, elle en reverse 98 % aux communes les attributions de compensation pour permettre aux communes et aux territoires de continuer à assurer les missions du quotidien. Les capacités financières réelles de la MGP sont donc dérisoires. Aujourd'hui, le changement se fait attendre. En juillet 2017, au Sénat, le Président de la République récemment élu, Emmanuel Macron, annonçait pourtant de futurs changements majeurs dans l'organisation du Grand Paris.

La fronde des départements contre la métropole " Macron " ». Novembre 2017 : « Métropole du Grand Paris : que va décider Emmanuel Macron ? » Janvier 2018 : « Quel sort Macron réserve-t-il à la métropole du Grand Paris ? » Octobre 2018 : « Métropolisation : le Paris en grand de Macron au point mort

Quel échelon supprimer ? Quel statut pour les territoires ? Quel périmètre pour définir la région capitale ? Qui doit exercer les compétences du quotidien ? Ces questions ne manqueront pas d'être évoquées ce soir. Si je devais résumer la situation, je citerais l'analyse de Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS : « Nous avons une métropole qui est tout à fait sous-calibrée, une gouvernance éclatée et une MGP croupion qui a quelques dizaines de millions d'euros de budget réel. Donc, il faut réformer et c'est un tel imbroglio qu'il faut réformer fort. Tout le monde le sait, mais personne n'est prêt à assumer les coûts politiques pour le faire.

car tout est exacerbé : les enjeux, les attentes, les ambitions et parfois, aussi, bien sûr, les déceptions. Pourtant, le contexte actuel est sans doute propice, comme le dit l'adage, à remettre le métier sur l'ouvrage. Je le disais récemment lors d'un colloque à l'Assemblée nationale consacré aux « métropoles résilientes » : la décennie 2010 aura été marquée par une relation passionnée, excessive même, avec le fait métropolitain et,, avec le Grand Paris. Elle s'est en effet ouverte, chacun s'en souvient, par une série de lois destinées à affirmer leur place sur la scène française et internationale loi relative au Grand Paris en 2010, la loi Maptam en 2014, la loi NOTRe en 2015. Elle s'est achevée dans un climat de méfiance ou de défiance, voire de rejet de ces mêmes métropoles, tour à tour accusées d'être responsables des fractures territoriales et invivables pour leurs habitants. Alors qu'une nouvelle décennie s'ouvre, tâchons, ensemble, d'y voir plus clair, au coeur de cette « assemblée des territoires ». Sur ce sujet, aucun consensus n'émerge, à l'exception d'un seul : la situation actuelle ne satisfait personne. La raison en est simple : elle ne permet pas au Grand Paris, en tant que réalité métropolitaine- non en tant qu'institution -d'être à la hauteur des immenses défis auxquels ce territoire doit répondre, aujourd'hui comme demain. Pour autant, je me permets de le rappeler, cette situation est le produit d'une histoire à laquelle nombre d'entre nous ont participé, une histoire faite de compromis, mais aussi d'occasions manquées et, il est vrai, d'un certain nombre de renoncements. Cette réalité, loin de la juger en procureurs implacables, nous devons la comprendre, pour éviter, collectivement, de refaire les mêmes erreurs. En effet, les destins de notre pays et du Grand Paris sont,, organiquement liés. Une large part de la capacité de notre pays à relever les immenses défis qui sont devant lui réside dans la réussite du Grand Paris. En cela, ce sujet relève, au sens le plus noble du terme, de l'intérêt général, transcendant nos personnes autant que nos mandats. Aussi, aujourd'hui, faisons en sorte d'examiner ce sujet avec des yeux à la fois informés par cette histoire et en même temps délestés, autant que faire se peut, des antagonismes et postures trop bien connus. Laissons, en somme, toute sa place à ce que Nietzsche, dans une jolie formule, appelait « l'innocence du devenir ». Comment, au fond, en sommes-nous arrivés à cette situation ?

Pour en sortir, faisons d'abord un rapide détour par l'histoire. Il n'est pas besoin de rappeler la place exorbitante qu'occupent Paris et sa région dans l'histoire et la géographie françaises. Elle est, à dire vrai, unique dans le monde. La complexité du paysage politique et institutionnel contemporain est l'héritière de cette histoire. La région Île-de-France, c'est en effet 1 300 communes, 11 établissements publics territoriaux, une métropole du Grand Paris, 8 départements, 800 syndicats, un conseil régional. La région Île-de-France, c'est également un État aménageur puissant, comme en témoigne la création de nombreuses opérations d'intérêt national, de villes nouvelles, ou de grandes infrastructures. Cette fragmentation institutionnelle se traduit logiquement, et malheureusement, par des politiques publiques elles aussi très fragmentées, évoquant une « orchestration sans chef d'orchestre », pour reprendre la belle formule du philosophe Wittgenstein. Cette situation, vous la connaissez et, comme moi, vous la déplorez. Pourtant, depuis les années 2000 et les actions de coopération engagées par Bertrand Delanoë entre Paris et certaines communes avoisinantes, depuis 2007, date du discours fondateur du président Sarkozy prononcé à Roissy, les réflexions n'ont pas manqué. Aussi, d'où viennent ces blocages et quels sont-ils ? Comme pour l'oeuf et la poule, il est difficile de faire la part des choses : sont-ce les fractures trop importantes qui empêchent l'émergence d'un destin commun ? Ou est-ce que l'absence d'un projet fédérateur conduit en retour à renforcer ces fractures ? Quoi qu'il en soit, le constat est là : le territoire grand-parisien concentre, de manière particulièrement exacerbée, l'ensemble des tensions et contradictions propres aux réalités métropolitaines. C'est une métropole-monde, dont le rayonnement ne se dément pas, mais c'est également un territoire marqué par de très grandes fractures, qui ne se résorbent pas.

que ces immenses disparités ont des conséquences très concrètes sur la qualité de vie des habitants, et logiquement, sur l'attractivité de la Tous ces constats nous ramènent au devenir de la région capitale, plus particulièrement à son devenir institutionnel. En tant que législateur, c'est ce qui vous intéresse au premier chef, et c'est bien normal,

durant tout le quinquennat, élus locaux et société civile ont également apporté leur contribution. Si je devais résumer ces propositions pour introduire notre débat, je je dirais qu'il existe trois grandes familles de scénarios, que je vais tâcher s'esquisser. Le premier privilégie l'échelle de la région, Le premier privilégie l'échelle de la région, prenant acte de la présence de nombreux sites essentiels à la vie de la métropole en grande couronne.

des élus communs aux échelons départementaux et régionaux et à assurer une rétribution des ressources financières. Enfin- c'est la troisième option -, on pourrait imaginer réunir les départements au sein d'un syndicat interdépartemental. La deuxième option privilégie le périmètre de la zone dense, c'est-à-dire, pour l'essentiel, de la petite couronne. Quant à la troisième option, je la développerai plus tard

M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite aborder le sujet par la face financière, si j'ose dire. La question du financement de la métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux a été repoussée depuis l'origine. Tout le monde convient que la formule choisie au départ tient davantage de l'usine à gaz que d'un financement clair des compétences exercées par chacun. Cette formule provisoire devait muter dans un second temps, mais le nouveau pacte financier a été différé. L'attribution de la cotisation foncière des entreprises, nous trouvons depuis lors, à chaque loi de finances, dans la situation d'arrêter le moins mauvais compromis possible pour parvenir à financer la mise en oeuvre des compétences des EPT et de la métropole, le tout en continuant à repousser la remise à plat de ce dispositif provisoire qui ne devait pas durer. durer. Évidemment, discuter du financement alors que la question des compétences et du périmètre reste pendante n'est pas simple. Toutefois, cette régulation annuelle n'offre pas de perspective claire pour les exécutifs et renforce la fragilité du système, alors même que le rôle de la métropole et des territoires est crucial pour la relance. donc la suivante, madame la ministre : ce mode de régulation du financement de la métropole et des territoires vous paraît-il soutenable, notamment compte tenu du contexte économique issu de la pandémie ?

Monsieur le sénateur, nous sommes d'accord sur le constat, à savoir que le schéma de financement de la MGP n'est pas viable à long terme. En effet, comme vous l'avez rappelé, l'organisation actuelle, malheureusement. Les règles actuelles sont illisibles, sauf pour quelques initiés, et les mécanismes de solidarité ne sont pas à la hauteur pour résorber les inégalités entre les territoires. Ce système vaut encore pour deux ans.

des difficultés existantes. Si la MGP ne produit pas suffisamment de services, c'est aussi parce qu'il a été décidé de ne pas lui transférer autant de compétences qu'à une autre métropole. Ensuite, les moyens financiers de la MGP sont très inférieurs à ceux d'une intercommunalité classique. Pour l'avenir, il faut donc prendre le débat par le bon bout en partant des objectifs avant de concevoir les bons tuyaux. L'objectif est, à mon sens, de construire un espace de solidarité, donc de partage des ressources financières entre territoires, c'est-à-dire entre collectivités, soit entre Paris et sa banlieue et entre l'est et l'ouest. On ne répondra pas aux enjeux de la région capitale en laissant chaque territoire replié dans son coin. À défaut d'une telle internalisation de la solidarité au sein d'une structure large, il faudra des transferts financiers plus directifs pour financer les grandes compétences structurantes. La parole est

Féraud. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la coopération entre la métropole, la ville de Paris et les communes qui sont incluses dans le périmètre de l'autoroute A86 a abouti à l'instauration d'une zone à faibles émissions, ou ZFE, métropolitaine au 1 juillet 2019. Poursuivant cette dynamique, le conseil métropolitain a adopté à l'unanimité la mise en oeuvre d'une nouvelle étape de la ZFE au 1 juin prochain, confirmant ainsi des objectifs ambitieux, parmi lesquels la restriction d'accès aux véhicules diesel en 2024. Néanmoins, pour assurer pleinement l'efficacité de cette ZFE, il faut aussi prévoir son contrôle et, pour cela, le système le plus performant est le contrôle-sanction automatisé.

Notons que celle-ci est à la seule charge des territoires et qu'elle requiert des investissements importants alors que le dispositif n'est que transitoire. Par ailleurs, son efficacité reste en pratique assez faible, puisqu'elle repose sur des contrôles aléatoires, véhicule par véhicule. Pour ces raisons, la vidéoverbalisation ne nous paraît pas être la bonne solution. Madame la ministre, ma question est la suivante : ne pensez-vous pas nécessaire et possible d'accélérer la mise en oeuvre par l'État des contrôles-sanctions automatisés pour permettre à la métropole d'exercer pleinement et sans attendre sa responsabilité en matière de réduction de la pollution ? La parole est est à Mme la ministre. Monsieur le sénateur, l'État s'est engagé activement dans la promotion des zones à faibles émissions, afin de diminuer la pollution dans les grandes agglomérations, et, ainsi, d'améliorer la qualité de l'air et donc les conditions de vie de nos concitoyens. La ville de Paris et la MGP se sont volontairement engagées rapidement dans la démarche, en prévoyant dès le 1 juin 2021 que les véhicules particuliers classés Crit'Air 4 et 5 et non classés ne pourront circuler en semaine de huit heures à vingt heures dans la ZFE. Concrètement, il s'agit de véhicules diesel immatriculés avant le 31 décembre 2005 et de véhicules à essence immatriculés avant le 31 décembre 1996. Cette interdiction sera étendue progressivement, comme prévu, aux autres vignettes. Dès juillet 2021, s'ajouteront les véhicules classés Crit'Air 3, et en janvier 2023, Crit'Air 2, afin d'atteindre l'objectif de 100 % de véhicules propres en circulation. Le ministère de la transition écologique avait missionné M. le préfet Bartolt en décembre 2018 pour préfigurer un système de contrôle-sanction automatisé, notamment pour les ZFE. Les conclusions de ces travaux ont été remises l'été dernier, et depuis lors, les administrations concernées poursuivent activement leurs travaux d'expertise, pour élaborer ce système de contrôle-sanction automatisé dans les meilleurs délais. D'ici à la fin de l'année, il devrait être possible de franchir une première étape en matière de contrôle du respect de la ZFE, en mettant en place un système de contrôle assisté par vidéo. Ce système de contrôle par des officiers de police judiciaire, avec l'assistance d'un système informatique et vidéo, permettra de réaliser effectivement des contrôles en attendant de pouvoir en réaliser un nombre plus important lorsque le système automatisé sera opérationnel.

la métropole actuelle ne fait absolument pas. Madame la ministre, quel est donc l'agenda du Gouvernement ? La parole est

Le deuxième privilégie le périmètre de la zone dense, c'est-à-dire pour l'essentiel de la petite couronne. Il existe enfin une troisième famille de scénarios, qui tous consistent à faire entrer les institutions de la région capitale dans le droit commun,

MGP serait alors réduite à un syndicat mixte de la zone dense réunissant autant que de besoin Paris, les EPT, les départements de la petite couronne et la région Île-de-France. C'est du moins et ces variantes sont présentés par leurs auteurs comme des étapes intermédiaires dans l'attente d'une réforme institutionnelle d'ampleur. Par nature, ils ne permettent donc pas d'embrasser l'intégralité des enjeux que je soulignais tout à l'heure.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ne suis pas un élu de l'Île-de-France ni un spécialiste du sujet.

les relations entre l'Île-de-France et les régions voisines. L'État est ainsi particulièrement vigilant à la bonne articulation entre régions.

Les projets autour de l'axe Seine pilotés par le préfet Philizot sont d'ailleurs emblématiques de cette approche intégrée

Il en est de même du projet de ligne nouvelle Paris-Normandie, la LNPN, conçue à la fois pour améliorer les liaisons des villes normandes vers Paris, mais aussi

la métropole du Grand Paris s'est donné comme objectif de contribuer à la réduction des inégalités territoriales, notamment en matière d'accès au logement. Au regard de la situation sociale dans laquelle nous nous trouvons, cet objectif est très loin d'être atteint. Les politiques publiques en faveur du logement social sont pourtant un levier essentiel dans la bataille contre les inégalités. C'est un enjeu majeur pour la MGP, puisque 72 % des demandes de logement social de la région sont localisées à l'intérieur de la métropole.

en permettant aux élus de provisionner les dépenses liées aux amendes, mais en faisant en sorte que la lutte contre les inégalités spatiales dans notre métropole du Grand Paris soit, enfin, à l'ordre du jour et une vraie priorité ? La parole est à Mme la ministre.

la production de logements sociaux relève essentiellement de la responsabilité des collectivités, qui fixent les objectifs dans le cadre de la planification et accompagnent les bailleurs par leur action en matière de foncier, d'urbanisme et de permis de construire. Il est vrai que les

depuis sa création, la métropole du Grand Paris soulève de nombreuses questions institutionnelles, juridiques et politiques, mais c'est bien le sens de la métropole du Grand Paris qui doit nous interroger ce soir. Conçue pour réduire les inégalités entre les habitants et améliorer leur cadre de vie, la métropole du Grand Paris se confrontera dès demain aux défis d'aujourd'hui : la démographie, la transition énergétique, la mobilité durable et l'attractivité économique. Néanmoins, ces défis ne pourront être relevés que si la population francilienne sait clairement à qui s'adresser pour telle ou telle situation. Soyons lucides : force est de constater que la métropole du Grand Paris est un objet politique peu identifié et peu connu. À ce jour, 208 conseillers et conseillères siègent au conseil métropolitain, pour y représenter les 131 communes membres. Je doute que les Franciliens concernés connaissent l'identité de leurs élus et le fonctionnement de ce conseil. Au millefeuille administratif français déjà encombrant s'est ajoutée la métropole du Grand Paris,

opaque : la première est une intercommunalité, certes débutante, mais souffrant encore de son image de colosse aux pieds d'argile ; la seconde, agile sur le plan des compétences et connue de tous, s'est au contraire imposée progressivement comme un échelon politique essentiel. Madame la ministre, ne doit-on pas travailler pour simplifier la question des objectifs, des moyens, des compétences et de leur leur périmètre, afin de dissocier distinctement la métropole du Grand Paris des autres collectivités et, ainsi, donner enfin corps à ce projet territorial, aujourd'hui en hibernation, dont nous attendons qu'il prenne son envol ?

Quelles que soient les solutions retenues, les intercommunalités procèdent toujours des communes, et c'est à l'échelon de ces dernières que se jouent les scrutins. Chacun a ainsi pu constater que la MGP et les programmes des EPT n'étaient pas au coeur des débats du scrutin municipal de 2020- c'est le moins que l'on puisse dire ! La légitimité d'une vaste intercommunalité pour trancher de grands enjeux stratégiques est, par nature, plus limitée que s'il s'agissait d'une collectivité à statut particulier. En effet, le conseil communautaire n'a pas été élu sur le fondement d'un programme électoral métropolitain clairement choisi par les électeurs. La seconde méthode, qui peut être complémentaire de la première, consiste à donner à une institution la possibilité de mettre en oeuvre un projet politique métropolitain clairement choisi par les électeurs c'est le modèle des collectivités à statut particulier, qui peuvent être dotées de compétences accrues par rapport aux collectivités de droit commun, voire issues de la fusion de deux échelons. Une collectivité est administrée par une assemblée élue au suffrage universel direct. Cette assemblée a sa propre légitimité dans l'hypothèse d'un scrutin de liste dans une circonscription unique. Elle peut se prévaloir de la claire validation par les électeurs du programme qu'elle met en oeuvre. Pour reprendre votre expression, monsieur le sénateur, les différents projets territoriaux portés par les diverses tendances politiques seraient périodiquement soumis aux électeurs qui choisiraient leur destin commun. Il faut cependant être clair : une telle collectivité ne ressemblerait en aucune manière à une métropole des maires, ou à une métropole à un autre échelon, ni à une communauté de départements. Elle serait, comme vous l'indiquez, dissociée des autres collectivités dans le respect du principe de non-tutelle.

la création de la métropole du Grand Paris avait déjà suscité de vifs débats sur la pertinence d'un nouvel échelon administratif et politique dans le millefeuille préexistant en Île-de-France. « La création de ce nouvel échelon devait d'ailleurs s'inscrire dans une réflexion nécessaire, plus globale, sur la répartition des compétences entre la région, la ville de Paris, les départements de la petite et de la grande couronne avec leurs spécificités, les nouvelles intercommunalités issues de la loi de modernisation En 2014-2016, de nombreux élus de terrain de tous bords politiques avaient aussi alerté sur le risque d'une relégation des territoires les plus éloignés du centre de Paris à la suite de la création d'une hyperstructure telle que la MGP. Malheureusement, ces préoccupations se confirment aujourd'hui, car le rapport de force institutionnel déséquilibré conforte les inégalités territoriales au sein de notre région. Cette problématique est particulièrement frappante dans le domaine des transports, quand les collectivités de Paris et de la petite couronne accaparent une part disproportionnée des investissements publics, alors que le réseau RER est au bord de l'implosion. Pour rappel, ce sont bien les habitants de la grande couronne qui ont besoin de transports en commun de qualité pour éviter de se déplacer en voiture et répondre à l'urgence environnementale. « Dans cette même logique, la création d'une zone à faible émission, décidée unilatéralement par la MGP pour limiter progressivement l'accès des véhicules

desserviront principalement la première couronne. Je crois que nous pouvons nous en féliciter, parce que le besoin était évidemment criant. Toutefois,

Je partage l'idée qu'il faut dépasser les clivages entre petite et grande couronne, zones denses et zones plus rurales. Tel est le sens des engagements de l'État, puisque, vous le savez, celui-ci s'est fortement engagé aux côtés de la région pour financer à hauteur de 1,4 2015-2020, le plan de mobilisation pour les transports. L'auteur du rapport insiste également sur le potentiel que représente l'aménagement des routes franciliennes, avec des voies réservées pour les transports en commun.

L'engagement de l'État pour l'amélioration des mobilités dans l'ensemble de l'Île-de-France se traduit également par la réunion, vendredi prochain, sur l'initiative du préfet de l'Île-de-France, d'une conférence stratégique sur les mobilités routières. La parole est à M. Pascal Savoldelli.

revanche, depuis sa création institutionnelle, nous traînons la question du statut de la métropole du Grand Paris : c'est un sujet et un enjeu politique et démocratique majeur, mais il est confisqué, détourné et instrumentalisé.

se trouvent en première ligne et ont une grande proximité avec nos concitoyens. Je pense en particulier aux communes, puisque ces dernières conservent la clause générale de compétence,

Madame la ministre, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais le mythe de l'utilité des fusions qui réduiraient les coûts a vraiment vécu. Si la métropolisation est une réalité que le redécoupage des régions a a favorisée et installée, le fossé créé entre cette institution et nos administrés renforce une crise démocratique déjà manifeste dans notre pays. Aux projets élaborés d'en haut, nous préférons fédérer de manière ascendante, en faisant de la réponse aux besoins l'ambition partagée de chaque échelon institutionnel.

que la logique d'investissement structurant à l'échelon de la région n'a pas suivi. Aujourd'hui, ces instruments ne sont plus dans l'air du temps, et les élus des territoires sont les plus légitimes pour faire des propositions. Néanmoins, on voit bien

faute de consensus sur la réforme institutionnelle, un outil assez souple qui nous permette de dégager quelques objectifs, un calendrier, des pistes de financement, et pourquoi pas un contrat régional régional d'intérêt national permettant de fédérer et de répondre aux attentes de nos concitoyens franciliens, et pas seulement en petite couronne, en matière d'investissements nécessaires à leur qualité de vie au quotidien ? La parole est à Mme la ministre. Monsieur le sénateur Arnaud de Belenet, je suis d'accord avec vous. Ce qui est essentiel, bien sûr, c'est de répondre aux besoins de nos concitoyens. Il faut éviter de nous perdre

comprend des territoires absolument stratégiques pour la vie de la métropole : Val d'Europe, Eurodisney, sites universitaires, etc. On voit bien

pour affirmer ici que la création de richesses, de valeur, d'emplois en Île-de-France et pour la métropole du Grand Paris peut passer par la grande couronne, grâce à quelques investissements. potentiels de développement en grande couronne, qui sont singuliers et nécessaires à la métropole urbaine et dense.

Pour compléter l'excellent exposé de ma collègue Lavarde, je dirai que, depuis que la V République existe, tous les Présidents de la République ont apporté leur contribution et une attention particulière à la région Île-de-France et à la capitale

sur la région capitale, sur le sort de Paris et sur tous les problèmes qui s'y posent ? Vous nous proposez des solutions, madame la ministre. En réalité, je plains votre situation, parce que nous avons compris que nous ne parlons pas de l'avenir de la métropole du Grand Paris. Vous évoquez trois solutions, autrement dit vous n'en avez aucune

À plusieurs reprises, un discours-programme nous a été annoncé et, à plusieurs reprises, il a été reporté. Puis, comme l'écrivait Louis XVI dans son journal à la date du 14 juillet 1789, rien En un sens, ne rien faire quand on ne sait que faire n'est pas la plus mauvaise option. En revanche, ne rien faire après avoir annoncé une réforme rapide et affirmer qu'un échelon du système territorial du Grand Paris devait disparaître, puis laisser entendre que cet échelon serait le département, et laisser penser que la région serait le bon échelon pour faire fonctionner tout en demandant à cette dernière de prendre davantage de responsabilités, notamment en matière de qualité de l'air, de lutte contre les inondations- c'est d'actualité ! -ou de relance économique constitue sans doute une très mauvaise option et traduit une pratique du pouvoir totalement délétère pour l'action publique. Pour agir, les institutions ont besoin de temps et de stabilité. Or, par votre volontarisme sans dessein et votre ardeur réformatrice dépourvue de contenu, vous avez mis la métropole du Grand Paris en attente ; vous l'avez enfoncée dans l'instabilité. Est-ce le bon jour ou le bon endroit pour réformer ? Peut-être le bon moment est-il passé ? Que faire en attendant ? « Allons-y », dit l'un et, finalement, il ne bouge pas. Comme l'a fait Beckett pour ces deux héros, nous pourrions ainsi résumer votre action pour la métropole du Grand Paris. Ce théâtre d'ombres serait comique s'il n'était joué au mépris des besoins des habitants de la région et du pays, dont la métropole est le coeur battant politique et économique. Les liens de la Seine-et-Marne et du Grand Paris ceux de l'ensemble de la grande couronne sont trop forts et trop essentiels pour que nous ne nous alarmions pas, au-delà des frontières de la métropole du Grand Paris, de cette situation préjudiciable au développement de toute la région et du pays. Alors que tous les acteurs s'accordent à dire qu'une réforme était nécessaire, vous n'avez pas su rassembler.

Pendant deux siècles, cela a plutôt bien fonctionné, jusqu'au jour où nos technocrates se sont emparés du problème et ont voulu le simplifier- doux euphémisme, puisqu'ils ont ajouté deux strates : l'intercommunalité et la métropolisation. Depuis lors, nous, les élus, déployons une énergie folle pour tenter de réduire ce millefeuille indigeste mes chers collègues, de ce que nous vivons en région Île-de-France : une ville-centre, Paris, ignorant les communes qui l'entourent ; une métropole qui prétend à des fonctions stratégiques, mais qui n'inclut pas le neuvième aéroport mondial, ni le plateau de Saclay, un des plus grands centres de recherche au monde ; à l'intérieur, des maires étouffant sous quatre couches d'administration et ayant perdu ce qui faisait le coeur de leur métier, à savoir répondre aux aspirations quotidiennes de leurs habitants. Aussi, madame la ministre, ne cherchez plus ! Je vous amène, avec humilité, la solution ! Ce qu'il faut faire, c'est supprimer une couche- rêvons un peu, deux couches -, pour redonner de l'air aux communes. Pour cela, on fusionnerait la métropole et la région en une région métropolitaine, qui conserverait toutes les fonctions stratégiques d'une métropole mondiale, avec, évidemment, schéma de cohérence pour les transports et compétences en matière

notamment l'aménagement urbain et l'urbanisme. Madame la ministre, ne pensez-vous pas que notre région capitale mérite d'accéder, enfin, au rang de grande métropole mondiale, en changeant de statut et de taille ? ailleurs, ne serait-il pas temps d'offrir aux maires de la première couronne un véritable choix d'organisation et la possibilité de retrouver une vraie liberté, au service de leurs administrés ? La parole

peut-être historique, de développer son rôle de métropole attractive et financière.

La complexité de la gouvernance de la métropole du Grand Paris contraste avec ses compétences limitées et exercées de manière croisée avec d'autres acteurs territoriaux, dont l'État. Son budget d'investissement- 50 millions d'euros -est lilliputien. Le périmètre territorial actuel, soit 7,3 millions d'habitants, ne correspond à aucune logique fonctionnelle. La métropole est un Grand Paris de l'État, non un Grand Paris des élus et des citoyens. Le déficit de légitimité démocratique et de notoriété auprès des citoyens a un effet dévastateur. Le dispositif ne répond ni à la diversité des territoires ni à leur identité, encore moins aux besoins de participation des élus et des habitants à la coconstruction des projets. Pourtant, jamais les enjeux n'ont été aussi importants ; jamais la complexité n'a été aussi forte. Il y a donc une immense contradiction qu'il faut résoudre, faute de quoi la première région européenne perdra des batailles au plan international et au plan local. local. Puisque vous êtes en responsabilité, madame la ministre, peut-on connaître votre position ? Voilà des lustres que l'on réfléchit à ces questions ... Faudra-t-il attendre la création d'un énième comité Théodule de Franciliens tirés au sort pour avoir la réponse ?

partons des projets, et réfléchissons ensuite à ce à quoi il semble le plus intelligent d'aboutir.

place. Les présidents de département défendent leur département, la présidente de région défend la région, les présidents des EPT défendent les EPT et les maires défendent les communes. Personne ne veut envisager de lâcher de bon coeur une partie de son pouvoir et, encore moins, de ses moyens. Là est le problème

Je m'inquiète de vous entendre dire qu'il faut reprendre les choses par le projet. Non, madame la ministre ! En matière d'inégalités territoriales, les écarts sont immenses ; la Seine-Saint-Denis s'enfonce

Merci,